Samedi 7 octobre, nous avons tous été meurtris par l’attaque terroriste islamiste du Hamas contre la population israélienne : des jeunes terminant un festival et des populations de kibboutz ont été sauvagement abattus, violentés, pris en otage. Nous avons basculé dans une inhumanité que nous pensions révolue. Nous pensons à tous les otages, dont nous demandons la libération. Depuis lors, l’escalade de la violence s’accélère. Les Palestiniens sont victimes de représailles ; des centaines de civils sont Hier, un hôpital a été bombardé, faisant des centaines de morts supplémentaires. Avec gravité, je veux dire ici que nous refusons de trier les morts civils. Le déplacement exigé par le gouvernement de Benyamin Netanyahou d’un million d’habitants de la bande de Gaza est intolérable et impossible. Il annonce un drame humanitaire sans précédent.

La France doit faire entendre sa voix dans le concert des nations. Elle doit affirmer haut et fort le respect des accords internationaux qui assoient la création de deux États, ainsi que la fin de l’occupation et de la colonisation. Madame la Première ministre, faisant nôtres les propos d’António Guterres, secrétaire général des Nations unies, nous exigeons un cessez le feu immédiat. La France va t elle porter à l’ONU une résolution en ce sens et faire reprendre à tous le chemin de la paix, si nécessaire à l’humanité ?

le 7 octobre dernier, une attaque terroriste sans précédent a touché Israël. Nous l’avons condamnée fermement, à plusieurs reprises – notamment avec vous, la semaine dernière. Au cours de cette attaque, vingt quatre de nos compatriotes ont perdu la vie. Sept sont encore portés disparus et plusieurs sont probablement retenus en otage à Gaza. face à l’horreur, Israël a le droit à la sécurité. Israël a le droit de se défendre dans le respect du droit international humanitaire. Comme l’a affirmé le Président de la République, rien ne justifie jamais que des civils soient pris pour cible. Aussi, à mon tour, permettez moi de dire mon effroi face à la frappe qui a touché l’hôpital al Ahli de Gaza, causant de nombreuses victimes palestiniennes. Je veux avoir une pensée pour les familles et les proches des victimes. Cela ne fait aucun doute, chaque vie compte. Les hôpitaux et le personnel médical sont protégés par le droit international humanitaire. Celui ci doit s’appliquer en toutes circonstances. Dès hier, le Président de la République a condamné très fermement cette attaque. Toute la lumière devra être faite sur ce drame. Les auteurs devront être identifiés et rendre des comptes. Madame la présidente Cukierman, dans ce contexte dramatique, la position de la France est très claire. Tout d’abord, nous sommes aux côtés de nos compatriotes. Je tiens à ce propos à saluer le travail de nos diplomates mobilisés jour et nuit.

Comme l’a déclaré le Président de la République hier, nous travaillons activement à leur libération. Plusieurs dizaines de nos concitoyens sont par ailleurs bloqués à Gaza, dans une situation extrêmement précaire. Nous les suivons individuellement et faisons notre maximum pour leur permettre de quitter ce territoire. Ensuite, je l’affirme de nouveau, les populations palestiniennes ne sont pas responsables de la situation. Nous avons annoncé un soutien supplémentaire de la France de 10 millions d’euros pour l’aide humanitaire à Gaza. Nous appelons à un accès humanitaire immédiat à Gaza, afin que l’aide des Nations unies puisse être acheminée et parvienne aux populations palestiniennes. C’est une urgence, des milliers de vies en dépendent. Enfin, du point de vue diplomatique, nous multiplions les contacts avec les pays de la région pour éviter l’escalade et un embrasement régional. Notre position est constante : une issue politique avec deux États vivant en paix et en sécurité. C’est le seul horizon pour la paix. Aux Nations unies, la France soutiendra cette après midi le projet de résolution présenté par le Brésil, qui condamne sans ambiguïté l’attaque terroriste tout en rappelant la nécessité de permettre l’accès de l’aide humanitaire et la protection de la population civile de Gaza. Madame la présidente Cukierman, la France cherchera toujours le chemin de la paix. Elle sera toujours une artisane de la sécurité et de la stabilité au Proche Orient.

par le meurtre de Dominique Bernard à Arras, ma ville, où l’émotion est à son comble. Une fois de plus, l’école est une cible pour ceux qui en veulent à nos valeurs, qui en veulent à notre République. le terroriste a trouvé sur son chemin des héros. Avec un sang froid admirable, enseignants, agents et policiers, au péril de leur propre vie, en ont sauvé de nombreuses. Les mots sont trop faibles pour les remercier et leur rendre hommage. Si le temps est au deuil et au recueillement, il n’occulte pas tout à fait celui des questions. Après trois décennies d’attentats et une trentaine de lois, l’arsenal juridique et policier existe. Est il suffisant ? L’attentat d’Arras montre malheureusement qu’il y a des failles. Pour autant, une énième loi de circonstance n’a guère d’intérêt. J’en appelle donc à la sagesse du Sénat pour trouver, dans la future loi Immigration, les réponses justes et fermes. Reste qu’il faut miser aussi et surtout sur une véritable politique éducative et parentale, impérative pour réarmer moralement la jeunesse. L’école doit demeurer un sanctuaire à l’abri de la violence de certains foyers et des idéologies mortifères, un lieu où l’on apprend et où l’on s’émancipe. Monsieur le ministre de l’éducation nationale, vous avez rencontré à Arras les enseignants, bouleversés par le drame. Ils attendent vos réponses à leurs questions. Pour ma part, je vous en pose deux. qu’allez vous faire, pour assurer la protection des établissements scolaires ? Les grilles et les circulaires ne suffiront pas ! Deuxièmement, qu’allez vous faire pour que le travail éducatif

cette exemplaire mobilisation dans des circonstances absolument terribles et dramatiques. Vous l’avez dit, Dominique Bernard est tombé en héros. Ses collègues qui sont intervenus sont des héros. sont des héros qui n’auraient pas dû l’être en de telles circonstances. La mission d’un enseignant, sa vocation, c’est de sauver des vies par la pédagogie, et non en s’interposant entre un terroriste armé et des élèves.

Des efforts et des progrès ont été réalisés ces dernières années, notamment depuis 2015, quand le gouvernement d’alors avait engagé un plan massif de sécurisation et des plans de mise à l’abri. Je le dis,

et de la jeunesse. Vendredi dernier, trois ans après l’assassinat de Samuel Paty, Dominique Bernard est mort poignardé devant son lycée. Lui aussi était professeur. Nos pensées vont à ses proches, ses élèves et ses collègues. C’est la richesse humaine qui fait toute la force de l’éducation nationale, mais elle s’amenuise. Au travers de nos enseignants, c’est le savoir et nos valeurs qui sont attaqués. L’école est en première ligne, mais elle ne peut être la seule réponse à cette violence qui trouve son lit dans l’effondrement de l’État social. de l’État social. L’école doit rester un lieu de transmission de savoirs et d’émancipation, un lieu où l’on apprend la tolérance et le vivre ensemble, un lieu où la communauté éducative se sent entendue. Malgré la sidération, la colère et la tristesse, il va de soi que l’école ne doit pas devenir une forteresse. Lundi dernier, une minute de silence a été observée dans tous les établissements scolaires. Hasard du calendrier, la commission d’enquête sur le signalement et le traitement des pressions, menaces et agressions dont les enseignants sont victimes reprenait ses travaux. À cette occasion, la faiblesse de la formation et de la préparation à la vie de classe des enseignants a été pointée du doigt. Il y a trois ans presque jour pour jour, monsieur le ministre, j’ai interpellé votre prédécesseur sur cette question. Rien n’a changé. On nous parle aujourd’hui d’un retour aux écoles normales, mais est ce vraiment le cap ? Hier, devant la commission d’enquête, la sœur de Samuel Paty nous a informés du défaut d’accompagnement institutionnel auquel s’était heurté son frère, alors qu’il cherchait soutien et protection avant son assassinat. appris que les dernières circulaires n’avaient apporté aucune amélioration dans la prise en compte de la parole des enseignants. Cette surdité institutionnelle est accablante. Au delà des discours de circonstance, nous attendons des actes et non des mots, monsieur le ministre. Quels seront les vôtres ?

Les islamistes veulent éloigner du savoir le plus grand nombre pour imposer leur obscurantisme. Notre école accueille tout le monde. Les islamistes veulent soumettre les femmes. Notre école accueille toutes les petites filles de France, avec tous les petits garçons de France. Les islamistes veulent imposer le règne de la religion. Notre école impose celui de la République et de la laïcité. Il est extrêmement important de réaffirmer ces enjeux. Madame la sénatrice, vous m’interrogez plus spécifiquement sur la question du respect de la laïcité à l’école et du soutien dû aux enseignants en la matière.

Je pense que nous, responsables politiques, avons aussi la responsabilité d’être unis derrière ces valeurs, notamment la défense de la laïcité dans notre école, et derrière les actes qui sont mis en place pour la faire respecter. Pour autant, nous n’avons évidemment pas épuisé le sujet. Vous l’avez dit, madame la sénatrice, il y a un enjeu de formation. formation initiale que nous sommes en train de refondre profondément, en lien avec les organisations syndicales représentatives des enseignants. J’aurai l’occasion de formuler des annonces dans les prochains mois sur ce sujet. Je pense aussi à la formation continue. Je le réaffirme ici,

pour les valeurs de notre école et de notre République, et j’espère pouvoir compter sur l’ensemble de la représentation nationale pour nous accompagner. La parole est à M. Jean François Rapin, pour le groupe Les Républicains.

Mais comment voulez vous que j’utilise des mots aujourd’hui pour exprimer l’impensable en perpétuelle répétition, l’impensable qui s’est reproduit à Arras la semaine dernière ? Tant de colère nous envahit tous, même si l’on doit rester digne – comme toujours en de telles circonstances… Cette dignité que l’on nous demande depuis toujours et à chaque fois ; cette retenue politiquement correcte dont nous sommes coupables après le père Hamel, après Nice, après, après le Bataclan et le Stade de France, après Samuel Patty et, aujourd’hui, après Dominique Bernard.

parce que, pendant des années, les ennemis de la France ont fait l’objet de trop de tolérance ? Face à ceux qui nuisent ou qui vont nuire à la France, nous ne pouvons plus montrer de faiblesse.

Monsieur le ministre, il ne faut pas se limiter à la surveillance. Il faut agir contre les ennemis de la République. À ceux qui n’aiment pas la France, je le dis : nous ne les retenons pas. Tout à fait ! Surtout, nous ne devons plus les attirer, ni en France ni en Europe, car, moi, la France, je l’aime La parole est à Mme Nadège Havet, pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants. Monsieur le ministre, dimanche à Arras, lundi dans toute la France, nous nous sommes rassemblés pour rendre hommage à Dominique Bernard, enseignant assassiné, trois ans après que l’a été Samuel Paty. Tous les deux ont été victimes de la barbarie, et celle ci porte un nom : le terrorisme islamiste. Nous témoignons notre soutien à sa famille, à ses collègues et à l’ensemble de la communauté éducative. Nous saluons le courage de celles et de ceux qui se sont interposés, ainsi que des forces de l’ordre qui sont intervenues rapidement. Nous pensons également aujourd’hui à nos amis belges et suédois, eux aussi endeuillés. Dominique Bernard est mort parce qu’il était un enseignant, un « porteur de flambeau », et parce que le djihadisme se projette contre l’école. Dominique Bernard est mort pour s’être interposé entre l’école, qui est au cœur de notre République et de sa promesse d’émancipation, et le fanatisme, dont l’objectif est exactement inverse. Après Arras comme après Conflans Sainte Honorine, il ne faut absolument pas tomber dans les pièges tendus par les défenseurs de cette idéologie mortifère, celle là même qui voudrait que nous fassions des amalgames ou que nous nous divisions. Il nous faut au contraire nous rassembler derrière nos valeurs communes, notamment la laïcité, et les réaffirmer. Je pense à Caroline Fourest, qui, avec d’autres, défend ce qu’elle nomme justement

La laïcité, c’est ce principe qui permet de croire ou de ne pas croire. Nous devons défendre ce cadre de neutralité et rappeler que, loin d’être la source de nos problèmes, il est au contraire la condition de notre vie collective. Monsieur le ministre, il est impératif que la parole puisse se libérer lorsque des propos se font menaçants. Comment mieux protéger nos enseignants tout en réaffirmant ce cadre qui nous est cher ?

Havet, vous avez raison : il faut que la parole soit libre. Pour que la parole soit libre, pour que les enseignants, les personnels de direction et l’ensemble des équipes éducatives

Nous en sommes à près de 360 signalements de contestation et de perturbation, qui s’apparentent parfois à des menaces de mort ou à l’apologie du terrorisme. Ce sont autant de signalements que j’ai adressés au procureur de la République, autant de procédures disciplinaires qui sont engagées. Pour les cas les plus graves plusieurs dizaines d’entre eux –, j’ai demandé aux chefs d’établissement l’exclusion de ces élèves sans délai, c’est à dire sans attendre la réunion des conseils de discipline. Si nous ne sommes pas fermes et clairs, nous n’arriverons pas à faire appliquer nos règles à l’école.

le souvenir de professeurs qui sont tombés pour l’école, on ne le piétine pas, on l’honore ; l’autorité de l’école et de la République, on ne la conteste pas, on s’y soumet.

Samuel Paty, Dominique Bernard : comment en sommes nous arrivés là ? L’école républicaine est en principe le lieu où chacun peut tirer le meilleur de lui même. L’école républicaine, c’est aussi le creuset de notre démocratie, le meilleur moyen d’intégrer et de souder notre communauté nationale. Or nous avons laissé le pacte se faire entamer et grignoter par petits bouts. En réalité, nous sommes aujourd’hui engagés dans un combat de valeurs : les valeurs républicaines contre l’intégrisme, les Lumières contre l’obscurantisme, la démocratie contre le fanatisme. Ce n’est pas un hasard si les professeurs d’histoire sont les premières cibles dans ce combat, si tous les enseignants sont en première ligne. Leurs témoignages se multiplient. Ils dénoncent les agressions verbales ou physiques, les intimidations qu’ils subissent au quotidien, encore amplifiées aujourd’hui par les réseaux sociaux et leur immédiateté. Au même titre que les élus, les professeurs sont les meilleurs garants de l’ordre républicain. Les enseignants doivent pouvoir transmettre nos valeurs communes en toute liberté. Pour leur permettre d’exercer leur métier, nous devons bien sûr assurer leur protection, mais cela ne suffira pas. Nous devons davantage valoriser leur rôle, peut être organiser les enseignements, notamment civiques, de façon à les laisser moins seuls dans l’accomplissement de leur mission et peut être intervenir dès leur formation pour mieux les préparer et leur permettre de continuer d’être ce qu’ils ont toujours été, les hussards de la République. Monsieur le ministre, l’heure est grave. Que comptez vous faire pour mieux protéger et mieux aider nos enseignants dans l’exercice de leur mission, qui est essentielle à notre démocratie ?

Alors que l’école devrait être, comme disait Jean Zay, « l’asile inviolable où les querelles des hommes ne pénètrent pas », un enseignant a une nouvelle fois été assassiné, au sein même de son établissement. Aujourd’hui se mêlent des sentiments de colère, de révolte et de sidération. Le groupe RDSE s’associe aux hommages rendus depuis vendredi dernier tombé parce que professeur, tombé parce que, comme l’aurait dit Jean Jaurès, il tenait entre ses mains « l’intelligence et l’âme des enfants ». Lieu d’instruction, d’inclusion et d’apprentissage de la liberté, notamment de conscience, l’école est devenue une cible. L’assaillant d’Arras a attaqué à dessein le symbole d’une République laïque, le lieu où se forme l’esprit critique, qui questionne les croyances et permet l’émancipation. Il a grandi en France et a été éduqué dans l’école de la République, là même où il a décidé de frapper. Au delà de l’obscurantisme et du fanatisme, ce drame doit nous interroger sur notre modèle républicain et sa pérennité. Lors d’une récente séance de questions au Gouvernement, je vous avais interrogé sur les réponses apportées à la banalisation de la violence du quotidien. prend ici une forme particulièrement horrifiante. Toutefois, comme en juin dernier, je veux vous parler de culture citoyenne et de solutions de moyen et de long terme pour soutenir les équipes éducatives, porter les valeurs républicaines et valoriser le sens de l’engagement dès le plus jeune âge. Je sais le Gouvernement attentif à ces sujets, comme en témoigne notamment le déploiement du service national universel (SNU). Vous nous trouverez à vos côtés dans ce combat. Le groupe RDSE défendra ainsi, dans quelques semaines, une proposition de loi, déposée par notre collègue Henri Cabanel, visant à renforcer la culture citoyenne. des propositions pour permettre à chacun de s’inscrire dans un projet commun, mais aussi de trouver son rôle et sa place dans une société apaisée. Monsieur le ministre, quels sont vos projets pour renforcer les outils d’éveil à la citoyenneté et favoriser le vivre ensemble ?

au terme de leur défilé, dans le cadre du débat démocratique qui fait l’identité et la grandeur de notre pays, les rues de la ville retentissaient des sirènes hurlantes des forces de police et de secours. À quelques dizaines de mètres, Dominique Bernard tombait sous les coups de couteau d’un individu animé par une idéologie terroriste islamiste. Arras, le Pas de Calais et la France entière étaient cruellement frappés par la barbarie, au cœur de la mission la plus noble de la République : l’éducation de ses enfants. L’horreur absolue s’abattait sur nous, nous replongeant dans les funèbres souvenirs des attentats de janvier et novembre 2015, faisant écho à l’assassinat de Samuel Paty, et nous rappelant qu’il est encore possible, en 2023, de mourir par le seul fait de transmettre le savoir. La République est en deuil. Je veux ici rendre hommage au courage de Dominique Bernard et saluer sa mémoire, assurer sa famille de notre soutien, former des vœux de rétablissement aux blessés et exprimer notre entière solidarité avec les élèves et les membres de la communauté éducative. Permettez moi également de saluer la réactivité et le courage de nos forces de sécurité et de nos services de secours. En ce temps de deuil, prenons la mesure de ce qui nous rassemble autour de ce que nous avons de plus cher, les valeurs de notre République : la liberté, l’égalité, la fraternité et la laïcité. Rappelons avec détermination que la République et la Nation doivent faire bloc face au fanatisme. Monsieur le ministre, vous avez établi un lien entre les événements qui se sont déroulés en Israël et cet attentat. Faisiez vous allusion au climat de haine et à l’effet de contagion suscités par ces événements ou avez vous connaissance d’une entreprise organisée et coordonnée, au delà des cellules terroristes familiales ou isolées, sur le territoire national ou en dehors de celui ci, qui viserait particulièrement notre pays ? d’alerte, nous sommes passés au niveau urgence attentat, pouvez vous nous éclairer sur la bonne manière de résoudre la redoutable équation qui permet de concilier la fermeté contre le terrorisme et le respect de l’État de droit, inventé par nos Lumières et marqueur des démocraties adultes telles que la nôtre ?

ont peur : la République les protège chaque jour et chaque nuit. La parole est à Mme Annick Petrus, pour le groupe Les Républicains. Monsieur le président, mes chers collègues, ma question s’adresse à M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse. Alors qu’un double hommage a été rendu aux professeurs Dominique Bernard et Samuel Paty, lâchement assassinés par des terroristes islamistes, islamistes, une rage sourde et une crainte certaine envahissent le monde enseignant. Comment peut on mourir d’enseigner en France en 2023 ? J’ai passé plus de trente cinq ans de ma vie à enseigner et j’étais heureuse de me rendre à mon établissement chaque matin. Aujourd’hui, cela ne serait certainement plus le cas. L’école est devenue la cible du terrorisme. Nous en avons la confirmation avec ces tragiques événements. À la colère et à la tristesse que nous éprouvons s’ajoute aussi l’effroi à l’idée que n’importe quel enseignant peut être aujourd’hui une cible. Dans une société de plus en plus violente, se retrouvent souvent bien seuls, face à des assaillants qui peuvent profiter d’un interclasse pour entrer tranquillement dans un établissement scolaire et tuer. Ils sont tout aussi démunis face à leur hiérarchie. Nos enseignants veulent un siècle de parole, non une minute de silence, le bras le long du corps, la montre en main. Ils veulent vivre pour enseigner, éduquer, instruire et élever : c’est leur mission et leur destin. Monsieur le ministre, nos enseignants attendent un soutien clair et sans faille de l’État. Aussi, quels moyens entendez vous mettre au service de nos établissements et de notre école, afin que celle ci puisse assurer sa mission essentielle, à savoir transmettre nos valeurs ? ailleurs, comment comptez vous réarmer nos enseignants et leur assurer une formation, à l’image de ce que furent les écoles normales à la fin du XIX siècle ? La parole

La parole est à Mme Monique Lubin, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Monsieur le ministre, je suis heureuse de vous entendre dire que les excédents de l’Agirc Arrco sont liés à des sacrifices qui ont été consentis par les salariés du secteur privé de notre pays

Les Républicains. Madame la Première ministre, votre gouvernement a publié hier les montants définitifs que percevront les collectivités territoriales au titre du filet de sécurité énergétique. Ce soutien de l’État était attendu, et je veux relayer ici les profondes inquiétudes des maires confrontés à l’explosion de leurs dépenses d’énergie, à l’inflation, à l’augmentation des charges de personnel, mais aussi à la remontée des taux d’emprunt.

puisque les critères de Bercy contraignent maintenant près de 3 500 collectivités territoriales à rembourser l’acompte perçu, alors qu’elles ont vu leurs dépenses exploser ! Dans mon département de Saône et Loire, près de deux communes sur trois ayant perçu un acompte vont devoir le rembourser. Dans ces conditions, madame la Première ministre, vous rendez vous compte que, après le piteux échec de vos contrats de confiance, ce dispositif est devenu le filet de la défiance entre l’État et les collectivités locales ?

Montchanin a reçu 374 000 euros et Montceau les Mines 275 000 euros. Le Gouvernement a appliqué les critères votés par le Parlement et a ventilé les crédits Finalement, monsieur le ministre, votre filet est à la sécurité ce que le match de dimanche fut à la Coupe du monde de rugby : un immense espoir devenu une terrible déception. Comme l’équipe de France, les collectivités locales ont joué le jeu, avec pugnacité, rigueur et engagement. Mais à la fin, c’est toujours Bercy qui gagne le match, en ne dépensant que 405 millions d’euros sur les 430 millions

aujourd’hui en attente d’un logement social, alors que 85 000 logements seulement seront mis en chantier cette année. Annoncées à cette occasion, les mesures du Gouvernement pour le logement vont dans le bon sens soutien à la transition écologique, bonification des prêts à la production et prorogation du prêt à taux zéro pour l’accession sociale. Toutefois, je ne vous apprends rien en vous disant que ces mesures ne permettront pas d’enrayer la crise profonde que nous traversons. Monsieur le ministre, l’histoire nous enseigne que l’État est massivement intervenu à chaque crise du logement : dans l’après guerre, dans les années 1950, dans les années 1970 1980 pour le logement social… Pourtant, aujourd’hui, votre gouvernement ne semble pas avoir pris la mesure de la situation. En témoigne le projet de loi de finances pour 2024 qui va nous être soumis. Répondre à la pénurie de logements sociaux, dynamiser le parc privé, loger nos étudiants, massifier la rénovation thermique, favoriser l’accession à la propriété, loger les plus fragiles… Jamais les enjeux n’ont été aussi nombreux. Ce que je vous demande aujourd’hui, ce que vous demandent les acteurs du logement, c’est un discours de vérité, un discours de clarté. Monsieur le ministre, face à toutes ces urgences, quelle est votre stratégie ? Quelles sont vos priorités ? Vous le savez,

ailleurs, comment expliquez vous le refus de la plainte du syndic ? Pour quelles raisons les arrestations sont elles intervenues seulement après la médiatisation de l’affaire ? La représentation nationale a pourtant voté, cette année, une loi permettant d’expulser plus rapidement les squatteurs. Monsieur le ministre, je sais l’immense travail fourni quotidiennement par les forces de l’ordre, mais des lacunes dans le traitement des plaintes font que les Français victimes de squats en sont réduits à recourir au tribunal médiatique pour faire avancer leurs dossiers. Que comptez vous donc faire pour remédier à cette situation, afin que les plaintes pour squat soient traitées rapidement et efficacement ?

toutes les situations de squat. Aux côtés des parlementaires, il s’est mobilisé pour simplifier et accélérer l’ensemble des mesures qui permettent de régler ces situations. Les moyens existent

d’amende. À cette occasion, un délit d’occupation frauduleuse des locaux à usages divers a élargi le spectre du squat aux autres types de locaux, en dehors du domicile. En la matière, les peines maximales ont été portées à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.

à quel point les finances locales étaient soumises à de fortes tensions budgétaires. Alors que les conseils municipaux s’apprêtent à voter avec grande difficulté leurs décisions budgétaires modificatives, les mauvaises nouvelles financières tombent de concert avec les feuilles automnales.

y découvrons que le nombre de bénéficiaires est encore plus faible que prévu. Pourtant, le comité des finances locales vous avait alerté quant aux difficultés opérationnelles à venir, qualifiant le dispositif de « trop peu, trop tard et trop compliqué

puisque vous aimez les métaphores, permettez moi de vous dire que ce filet est davantage un filet de pêche qui visait à draguer les communes et que les mailles étaient si larges qu’une grande partie des collectivités s’en sont trouvées exclues

ce plan se termine à la fin de l’année en cours, votre décision d’arrêter le versement des aides au 15 octobre dernier, afin d’éviter les retards de paiement, a provoqué une légitime levée de boucliers des professionnels, le gazole, principal poste de charge des pêcheurs, n’ayant cessé d’augmenter en 2023.

Par ailleurs, vous annoncez, pour 2024, un accord avec le groupe Total Énergies au sujet de la mise en place d’une ristourne de 13 centimes d’euros à la charge du pétrolier, dans le cadre de l’introduction de biocarburant dans le gazole.

et après le plan de sortie de flotte post Brexit, qui a amputé notre capacité de production de manière significative, le moment est venu de faire entendre la voix de la France à Bruxelles auprès de nos partenaires européens. La situation est grave ! Voulons nous la mort de la pêche française ? Une telle disparition nous obligerait à importer encore davantage de produits de la mer de pays tiers qui ne respectent aucune de nos normes environnementales et sanitaires. Monsieur le secrétaire d’État, notre modèle de pêche français doit être sauvé

Afin de porter la part d’énergies renouvelables dans notre consommation finale d’énergie à 33 % d’ici à 2030, ce texte permet aux communes de définir les zones d’accélération dans lesquelles elles souhaitent prioritairement voir s’implanter des projets d’énergies renouvelables. À la suite d’une réunion organisée récemment dans le département du Doubs, en présence des élus locaux, des services de l’État et des principaux acteurs du marché de l’énergie, de nombreuses questions sont remontées sur les difficultés d’application de cette disposition. ne sont pas propres à ce territoire, comme en témoignent les expériences similaires vécues par plusieurs de mes collègues. Comme vous le savez, les élus doivent rendre leurs propositions avant le 31 décembre 2023.

Aussi, je souhaiterais savoir comment le Gouvernement entend répondre aux inquiétudes des élus locaux sur la mise en place des ZAER dans le délai imparti. Quand les décrets d’application tant attendus dans nos territoires

des énergies renouvelables, nous avons décidé, ensemble, de mettre les élus locaux au cœur du processus de planification énergétique. C’est un gage de réussite de la planification écologique voulue par le Président de la République et par la Première ministre. Concrètement, la loi précise que les maires ont désormais la possibilité de définir des zones d’accélération, dans lesquelles ils souhaitent que soient développées des énergies renouvelables,

Mes chers collègues, par lettre en date de ce jour, le Gouvernement demande l’inscription à l’ordre du jour du mardi 24 octobre, l’après midi, d’une déclaration, suivie d’un débat, en application de l’article 50 1 de la Constitution, relative à la situation au Proche Orient.

14 minutes pour le groupe Les Républicains, 12 minutes pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, 10 minutes pour le groupe Union Centriste, 8 minutes pour les autres groupes, 3 minutes pour un sénateur non inscrit.

observations ?… Il en est ainsi décidé. Par ailleurs, le Gouvernement demande le retrait de l’ordre du jour des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique, qui étaient inscrites le mercredi 8 novembre

le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur le projet de loi pour le plein emploi ont été publiées.